La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 14 mars 2024 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n’y a pas d’observation ?… Le procès verbal est adopté. En application de l’article 32 de l’ordonnance n° 58 1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, M. le président du Sénat a reçu de M. le ministre de l’intérieur et des outre mer une communication de laquelle il résulte que, à la suite des opérations électorales du dimanche 17 mars 2024, Mme Marie Jeanne Bellamy a été proclamée sénatrice de la Vienne. Son mandat a débuté ce lundi 18 mars à zéro heure. Au nom du Sénat tout entier, je souhaite à notre nouvelle collègue la plus cordiale bienvenue. j’ai le regret de vous faire part du décès de nos anciens collègues Louis Minetti, qui fut sénateur des Bouches du Rhône de 1978 à 1998, et Jacques Donnay, qui fut sénateur du Nord de 1999 à 2001. Mes chers collègues, par lettre en date du vendredi 15 mars, la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport demande au Sénat, en application de l’article 5 de l’ordonnance n° 58 1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, de lui conférer les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête, pour une durée de six mois, afin de mener sa mission d’information sur les modalités de constitution d’une société commerciale par la Ligue de football professionnel en application des articles L. 333 1 et suivants du code du sport introduits par la loi n° 2022 visant à démocratiser le sport en France. La conférence des présidents examinera cette demande lors de sa réunion de demain, mercredi 20 mars.

mer. Madame la ministre, je souhaitais attirer l’attention de M. le ministre de l’intérieur et des outre mer sur les financements octroyés à la Tunisie. Dès le début de l’année 2023, alors que notre assemblée commençait ses travaux sur le projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, le président tunisien déclarait dans un communiqué qu’« il existe un plan criminel pour changer la composition du paysage démographique en Tunisie », relayant la théorie complotiste trop répandue du grand remplacement. Lors d’un conseil de sécurité nationale convoqué sur le sujet, il avait même évoqué des « hordes de migrants clandestins », dont la présence en Tunisie serait, selon lui, source de « violence, de crimes et d’actes inacceptables

Depuis lors, la Tunisie a mené des campagnes massives d’arrestation et d’expulsion de migrants, notamment depuis la ville de Sfax, point de départ de personnes migrantes vers l’Europe. Ces migrants sont emmenés par des forces de police vers la région frontalière avec la Libye et l’Algérie ; ils y sont abandonnés dans des zones désertiques, sans eau ni nourriture ; ils y subissent la chaleur et y ont trop souvent trouvé la mort. Nous sommes profondément préoccupés par l’expulsion de migrants, réfugiés et demandeurs d’asile de Tunisie vers les frontières avec la Libye, et aussi avec l’Algérie », avait déclaré le porte parole adjoint du secrétaire général des Nations unies à l’été 2023. Ces épisodes ignobles suscitent des interrogations sur le financement annoncé par le ministre de l’intérieur. Aussi, je souhaiterais connaître le cadre précis de ce financement destiné, selon lui, à permettre d’« acquérir des équipements nécessaires et organiser les formations utiles, notamment des policiers et gardes frontières tunisiens », pour « contenir le flux irrégulier de migrants » et « favoriser le retour de ces migrants Aucune aide ne peut être octroyée sans contrôle, d’autant que la Tunisie a récemment interdit la venue d’une mission parlementaire du Parlement européen. Je voudrais donc connaître le cadre légal de cet accord bilatéral de financement, le calendrier de ce financement, la nature des équipements qui ont pu être acquis grâce à cette aide de notre pays, le type de formations qui auraient été dispensées dans ce cadre ; surtout,

constituent un défi majeur pour la Tunisie, à laquelle la France tient à assurer sa solidarité et son soutien dans les efforts qu’elle déploie pour gérer ces flux et renforcer la stabilité régionale. L’objectif du Gouvernement est de prévenir ce phénomène migratoire en fournissant l’acquisition d’équipements nécessaires, ainsi qu’en organisant des formations ciblées, notamment au profit des policiers et gardes frontières tunisiens, afin de contribuer à la maîtrise des flux irréguliers de migrants et de favoriser leur retour dans leur pays d’origine. À ce titre, une convention entre Civipol, opérateur du ministère de l’intérieur et des outre mer, et le ministère de l’intérieur tunisien a été signée le 13 décembre 2023, de même qu’un contrat entre Civipol et Idemia, expert mondial des systèmes biométriques de sécurité, ayant pour objet la mise à niveau du système biométrique et le renforcement de la police technique et scientifique tunisienne. Cette opération, dont le coût global s’élève à 8,9 millions d’euros, monsieur le sénateur, est financée à hauteur de 5 millions d’euros par la France. Elle couvre la livraison de matériels et de licences, ainsi qu’un service de maintenance assuré jusqu’en 2025. Le parc d’équipements mobiles sera également élargi ; il comprendra le renouvellement des huit stations d’identification dans les consulats tunisiens en France, favorisant l’identification accélérée des Tunisiens à l’étranger.

et des outre mer. Madame la ministre, l’Italie communique chaque jour les données relatives aux entrées d’immigrés clandestins sur son sol et en fournit chaque mois un tableau de bord complet, depuis 2017. La France est beaucoup moins transparente en la matière. Ce que nous savons, c’est que, après une légère baisse liée à la crise sanitaire, les arrivées de mineurs non accompagnés (MNA) se sont multipliées en 2023, notamment après la crise de Lampedusa en Italie. Leur nombre a été multiplié par quatre entre 2014 et 2023, passant de 5 033 à 19 370

comme vous le savez, les mineurs non accompagnés, âgés de moins de 18 ans et séparés de leurs représentants légaux sur le sol français, relèvent de la compétence de plusieurs ministères, mais aussi de celle des départements, au titre de l’aide sociale à l’enfance. Le ministère de l’intérieur et des outre mer apporte un soutien à ces derniers dans la phase d’évaluation de la minorité, rendue spécialement difficile en raison de l’absence de documents d’identité ou des lacunes de l’état civil des pays d’origine. L’étranger reconnu MNA bénéficie sur le territoire d’une protection absolue à l’encontre de tout éloignement forcé durant sa minorité.

64,3 % d’Asie – à 60,7 % d’Afghanistan – et 31,8 % d’Afrique. Le taux des protections reconnues par l’Ofpra aux MNA demeure élevé – 82,5 % –, à l’instar des années précédentes, et excède nettement le taux global de protection de l’Office, qui est de 29,2 %. reconnu réfugié ou bénéficiant de la protection subsidiaire peut demander la réunification familiale pour ses père et mère, accompagnés éventuellement par ses frères et sœurs mineurs non mariés. Cette procédure est une voie d’immigration fondée, rigoureusement appliquée, en particulier pour ce qui concerne la documentation et la réalité des liens familiaux. Le ministère de l’intérieur et des outre mer cherche bien à détecter, le plus en amont possible, les ressortissants

mer. Madame la ministre, au mois de mai 2018, à l’occasion du Congrès des maires de France, Emmanuel Macron avait dit souhaiter que les préfets puissent échanger avec les maires sur la présence, dans leurs communes, des personnes fichées pour radicalisation islamiste identifiées comme les plus à risque, qui sont recensées dans le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT). Cette annonce présidentielle avait été suivie par la circulaire du 13 novembre 2018, qui confiait aux préfets la tâche de transmettre toutes les informations nécessaires aux maires maires afin d’améliorer la protection des Français, notamment dans le cadre de la radicalisation violente de personnes présentes dans leurs communes. Malheureusement, la circulaire n’a produit aucun effet sur le terrain, et il a fallu attendre le tragique attentat du lycée d’Arras, à l’automne 2023, perpétré par un énième individu fiché S, pour que ce sujet soit de nouveau mis sur la table

Vous le voyez, madame la ministre, lorsqu’il s’agit de la sécurité des Français, les clivages s’effacent au bénéfice du bon sens : l’échelon municipal doit prendre toute sa place dans la protection de nos concitoyens.

Mme la ministre déléguée. Monsieur le sénateur Durox, les fiches S constituent un outil de renseignement permettant une mise en attention et une surveillance discrète des individus par les services de renseignement.

afin de ne pas contrarier la discrétion s’attachant à cette surveillance ni de risquer de compromettre des enquêtes en cours. C’est pourquoi le Gouvernement n’est pas favorable à l’ouverture de l’accès aux fiches S du fichier des personnes recherchées (FPR) aux maires des communes dans lesquelles résident les personnes concernées. a cependant souhaité faire en sorte que les maires soient pleinement associés aux dispositifs de prévention et de prise en charge de la radicalisation mis en œuvre par les services déconcentrés de l’État. Au demeurant, il s’est toujours pleinement engagé en faveur du renforcement de l’information des maires, pour la protection de nos concitoyens.

par les agents de police municipale, en application de l’article 21 2 du code de procédure pénale. Par ailleurs, depuis la circulaire du ministre de l’intérieur du 13 novembre 2018, les préfets sont autorisés à partager certaines de ces informations confidentielles et nominatives avec les maires et présidents d’intercommunalités, dans le cadre des groupes restreints des conseils locaux ou intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance, sous réserve de l’accord du chef du service de police et du procureur de la République territorialement compétents. Enfin, la question de l’ouverture d’un accès partiel et proportionné des maires à d’autres fiches du FPR fait actuellement l’objet d’un examen approfondi par les services du ministère de l’intérieur et des outre mer, étant observé que les policiers municipaux disposent, depuis plusieurs années, d’un accès de plus en plus étendu aux fichiers relevant de l’État, pour leur permettre de traiter les infractions relatives à la sécurité qu’ils sont habilités à constater. Le Gouvernement entend poursuivre cette dynamique, en élargissant l’accès des policiers municipaux à d’autres fichiers du ministère de l’intérieur et des outre mer. Ce sujet pourra faire l’objet de discussions à l’occasion du Beauvau de la police municipale.

Le Gouvernement a fait montre à plusieurs reprises de son incapacité à expulser les fichés S, qui représentent pourtant un grave danger pour nos compatriotes. De même, les filières d’immigration légale et illégale charriant une partie de ces fichés S ne sont pas non plus taries, en dépit des rodomontades de M. Darmanin. Vous êtes visiblement dépassés par la situation. Aussi, permettez aux maires de France, qui le demandent, de protéger les Français

Malgré la prévention assurée par les services de l’État, nous assistons à une recrudescence de ces actes frauduleux. Il serait aujourd’hui possible de minimiser la portée de ces pratiques en permettant aux contribuables de consulter l’état de leurs contraventions sur le site des immatriculations et, ainsi, de vérifier l’authenticité de la de la demande de paiement. Madame la ministre, j’aimerais donc savoir si vous envisagez de permettre aux Français d’accéder à la consultation de leurs contraventions sur le site des immatriculations ou par un autre moyen sur Pouvez vous également me faire état des moyens mis à la disposition des forces de police et de gendarmerie pour lutter contre cette fraude en ligne et mieux en protéger nos concitoyens et nos services publics ? La parole est à Mme la ministre

Plus de 110 000 appels et quelque 10 000 courriels ont été traités à ce titre. Enfin, sachez qu’il est déjà possible de consulter ses contraventions sur le site de l’Antai, le parcours « Consulter mon dossier d’infraction ». Par ailleurs, les moyens cyber de la police et de la gendarmerie montent en puissance : en témoigne la création d’une agence du numérique des forces de sécurité intérieure, du commandement du ministère de l’intérieur dans le cyberespace, ainsi que de l’office anti cybercriminalité de la direction nationale de la police judiciaire.

de mieux orienter les particuliers victimes de cyberdélinquance. Vous pouvez compter sur la détermination du ministre de l’intérieur à renforcer l’ordre public dans l’espace numérique, ainsi que la protection de nos concitoyens, de nos entreprises, de nos collectivités et de nos administrations sur internet. Nous savons, madame la sénatrice, que nous pouvons compter sur vous dans ce combat. La

assimilant les sapeurs pompiers volontaires à des travailleurs. Les membres de ce comité estiment que les sapeurs pompiers volontaires subissent un traitement discriminatoire en matière d’indemnisation et de temps de travail. Ils condamnent également l’implication de sapeurs pompiers âgés de 16 ans à 18 ans dans des opérations de lutte contre l’incendie. Si cette décision n’a pas de force contraignante, elle remet en revanche fondamentalement en cause notre modèle de sécurité civile, qui, je le rappelle, repose essentiellement sur le volontariat. Dans le même temps, le rapport commandé l’année dernière par le ministre de l’intérieur à l’inspection générale de l’administration plaide également pour une révision des contraintes qui pèsent sur les sapeurs pompiers volontaires et formule diverses propositions.

Vous avez raison de le souligner, la complémentarité fait la force de la sécurité civile en France, qu’il s’agisse des actions complémentaires de l’État, des collectivités et des associations, ou encore de la complémentarité entre les sapeurs pompiers professionnels et les sapeurs pompiers volontaires. Depuis de nombreuses années, le Gouvernement et le Parlement ont veillé à mettre en place des mesures destinées à conforter la spécificité des sapeurs pompiers volontaires français, caractérisés par leur engagement citoyen au service de nos concitoyens, notamment le principe selon lequel cet engagement ne peut être assimilé à celui d’un travailleur.

Le modèle français de sécurité civile repose sur l’engagement quotidien de 253 000 sapeurs pompiers, civils et militaires, en particulier sur celui de 198 700 sapeurs pompiers volontaires. Ces derniers incarnent la richesse et la complémentarité des forces qui, chaque jour, assurent la protection de nos concitoyens. objectif est bien de protéger l’engagement volontaire et citoyen au sein des services d’incendie et de secours. Enfin, le ministre de l’intérieur et des outre mer a annoncé la tenue d’une grande concertation portant sur notre modèle de sécurité civile, dans le cadre d’un « Beauvau de la sécurité civile » ; nous

sur le modèle français de sécurité civile, en particulier sur l’organisation de nos services départementaux d’incendie et de secours. Je voudrais à mon tour saluer le courage, l’engagement et le dévouement

Inédite dans son principe et par son ampleur, cette campagne de vaccination vise à mieux protéger la santé des animaux et celle des hommes. À l’échelle internationale, la France est le premier grand pays exportateur de volailles à déployer un tel dispositif innovant pour renforcer la protection des élevages. À la mi mars 2024, plus de 22 millions de canards ont fait l’objet d’une vaccination obligatoire contre l’IAHP pour l’ensemble des élevages de plus de 250 canards dont les produits sont commercialisés sur tout le territoire métropolitain. Cette campagne vaccinale, dont le montant avoisine les 100 millions d’euros, est financée à 85 % par l’État pour les deux premières doses et à 100 % pour la troisième dose. Les modalités de financement de la prochaine campagne vaccinale seront définies dans les semaines à venir, en concertation avec les filières professionnelles.

preuve de l’efficacité du dispositif. Seuls dix foyers sont aujourd’hui recensés, contre trois cent quinze à la même date l’an passé. La situation sanitaire favorable a d’ailleurs conduit le ministère à abaisser le risque influenza aviaire à « niveau modéré

prévues par l’arrêté du 24 mars 2017, qui fixe les conditions d’accueil et de prise en charge des animaux importés saisis dont le statut sanitaire est incertain. Cet arrêté détermine que tous les points d’entrée du territoire français disposent d’installations et d’équipements nécessaires pour l’hébergement temporaire et l’isolement de ces animaux. Une station animalière doit notamment disposer d’un local sécurisé, facile à nettoyer et à désinfecter, doté de cages ou autres équipements adaptés pour l’accueil de petits mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons et invertébrés, en vue de les nourrir et de leur administrer les soins minimums, dans l’attente d’une décision administrative et de leur placement dans une structure d’accueil pérenne. Aujourd’hui, force est de constater que de telles structures existent seulement au sein de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle et dans le port de Calais. Par exemple, les services des douanes de Roissy ont encore récemment saisi une vingtaine de scorpions, qui étaient placés dans des boîtes. L’existence d’une station animalière a permis de sécuriser la détention de ces animaux, avant qu’ils ne soient placés. Le reste des points d’entrée du territoire ne bénéficiant pas de ce type de locaux, où sont hébergés ces animaux ? Dans la majorité des cas, ils seraient stockés dans les locaux des services des douanes, ce qui pose un problème en matière tant de contrôle des risques sanitaires que de sécurité pour ces animaux, pour le personnel et pour les voyageurs.

Dans les points d’entrée des voyageurs, les contrôles sanitaires sur les animaux de compagnie en provenance des pays tiers à l’Union européenne sont réalisés par les agents de la douane. Ces derniers sont également susceptibles d’identifier des introductions frauduleuses d’animaux non déclarés – vous venez d’en donner un exemple –, lors de contrôles sur des bagages ou marchandises de fret en provenance des pays tiers. La gestion de ces animaux au statut sanitaire incertain doit être effectuée dans le respect des réglementations applicables en matière de santé et de bien être animal, et de protection des espèces menacées d’extinction. C’est dans cette approche « Une seule santé » que l’arrêté du 24 mars 2017 a requis, à la suite de plusieurs cas d’interceptions à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, la mise en place d’une solution d’hébergement et d’isolement dédiée, pour organiser la prise en charge de ces animaux dans les points d’entrée désignés. L’objectif général de cet arrêté est de mettre à disposition des agents de la douane une structure d’isolement permettant d’héberger temporairement un animal non conforme saisi, afin de pouvoir gérer sereinement la prise de décision concertée avec les services chargés des contrôles vétérinaires sur le devenir à long terme de l’animal. Cet arrêté prévoit également la possibilité pour les points d’entrée de conventionner avec un prestataire, modalité que plusieurs points d’entrée mobilisent avec succès. L’infrastructure mise en place au sein de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, principale porte d’entrée identifiée du trafic illicite d’animaux, a déjà permis à plusieurs reprises d’héberger des animaux interceptés sur les plateformes aéroportuaires parisiennes. Il convient de souligner que cette infrastructure est mutualisée et permet

si l’on peut se réjouir de l’organisation des championnats du monde de cyclisme sur route en Haute Savoie en 2027, la violence des propos de M. Michel Callot, président de la Fédération française de cyclisme, et de M. David Lappartient, président de l’Union cycliste internationale, à l’égard des parlementaires opposés opposés au vélodrome surprend, surtout lorsque l’on sait que les seuls droits d’organisation de cette compétition s’élèvent à 18 millions de francs suisses. Le montant de l’indemnisation de la construction du vélodrome abandonné

et parties prenantes ». Malgré nos nombreuses relances, rien de tel n’a jamais été organisé. Il serait bon dans ce pays que les instructions formelles des ministres se traduisent réellement dans les faits. Quinze mois plus tard, il n’est jamais trop tard ! La parole est est à Mme la secrétaire d’État. Monsieur le sénateur Loïc Hervé, vous avez voulu alerter la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques sur le projet de construction d’un complexe sportif

Le 7 février dernier, le conseil municipal de La Roche sur Foron s’est prononcé contre la vente du terrain qui devait permettre la construction du complexe sportif, notamment le vélodrome. Le ministère des Sports et des jeux Olympiques et Paralympiques a pris acte de la décision du conseil municipal.

qui sera une occasion supplémentaire de mettre en valeur votre région. Comme il s’y est engagé par un courrier en date du 16 février 2024, le préfet de Haute Savoie organisera dans les prochaines semaines une réunion avec l’ensemble des élus du territoire à ce sujet. La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques reste extrêmement vigilante sur les modalités de gouvernance de l’organisation, qui reste à l’initiative du conseil départemental et de la Fédération française de cyclisme. Mme Amélie Oudéa Castéra veillera ainsi à ce que l’ensemble des acteurs du territoire,

L’Agence nationale pour l’information sur le logement (Anil) a publié la carte des loyers 2023. Le constat est frappant : plus l’on s’approche du Luxembourg, plus le loyer est élevé. Nombre de communes du nord de la Meurthe et Moselle, département dont je suis élue, et de la Moselle se situent dans la tranche la plus élevée des loyers en France, au delà de 12 euros le mètre carré. s’ajoute l’augmentation du coût de l’énergie et du transport, alors que les transports en commun bénéficient davantage aux déplacements transfrontaliers qu’aux déplacements interurbains, notamment grâce à la mise à disposition gratuite de cars par le Luxembourg. Pour répondre aux mêmes problèmes d’attractivité, l’État attribue une prime aux fonctionnaires résidant dans 133 communes proches de la Suisse, si vous voyez ce que je veux dire… Oh oui ! Cette prime de résidence, d’un montant équivalent à 3 % du traitement indiciaire, vise à aider les fonctionnaires à se loger loger et à rester. Si cette mesure fait sens dans les territoires frontaliers à la Suisse, elle le fait tout autant pour les territoires frontaliers au Luxembourg, qui font face aux mêmes défis et aux mêmes difficultés. Par conséquent, madame la secrétaire d’État, je souhaite avoir l’avis du Gouvernement sur cette proposition.

au regard de l’action menée dans l’Ain et en Haute Savoie. En portant la création d’une indemnité de résidence spécifique aux communes situées dans l’aire d’attraction du bassin genevois, le Gouvernement a apporté une réponse à une situation d’urgence, face à la baisse d’attractivité des emplois publics de ces territoires. De fait, la fixation des critères devant être aussi objective que possible et orientée d’abord sur le coût du logement, cette nouvelle indemnité repose sur le zonage prévu par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi Alur, qui classe les communes selon le degré de tension sur le marché locatif local. Elle bénéficie aux agents des communes classées en zone de forte tension, dite zone A, qu’à leurs communes limitrophes appartenant à la même unité urbaine, et représente 3 % du traitement de base. Une généralisation de cette indemnité de résidence spécifique à l’ensemble des grandes métropoles ou zones transfrontalières qui ne seraient actuellement pas éligibles à l’indemnité de résidence de droit commun n’est pas une réponse adaptée aux problématiques particulières d’attractivité que connaissent certains employeurs. Celles ci concernent davantage des métiers et des conditions d’exercice spécifiques et appellent des réponses structurelles, qui figureront dans le projet de loi que mon collègue

Le groupe dispose de deux sites industriels situés respectivement à Amiens, en Picardie, et à Carling, en Moselle. Le site d’Amiens est le seul site européen de production d’acides aminés biosourcés à destination de la nutrition animale. Metex entend se positionner sur trois chantiers, à savoir produire, commander et acheter en France, afin de participer à notre souveraineté alimentaire.

En 2024, le prix du sucre, de 30 % supérieur au prix de référence, les importations chinoises hors règles internationales de concurrence commerciale et les droits de douane prohibitifs pèsent dangereusement sur la compétitivité du site amiénois, qui rencontre de grandes difficultés. La production d’acides aminés notamment destinés à nos élevages exige le rétablissement d’une concurrence loyale. Je rappelle que la lysine est importée en Europe sans droit de douane et sans tenir compte du bilan carbone, dont l’économie, s’il fallait compenser la production par du soja à hauteur de 50 %, est estimée à 6 millions de tonnes pour l’empreinte carbone

en Europe. Il s’agit d’un fournisseur important de nos éleveurs et de notre industrie pharmaceutique. Qui plus est, elle contribue à leur décarbonation. Malheureusement, le processus d’adossement à un nouvel acteur industriel lancé par le groupe il y a quelques mois afin de pérenniser son activité et de financer son développement n’a, à cette date, pas permis d’aboutir à une solution satisfaisante. Le groupe a donc sollicité l’ouverture de procédures collectives, afin de poursuivre cette recherche dans un cadre adapté et sécurisé. Les prochains mois pourront ainsi être utilisés pour rechercher de nouveaux partenaires à même de reprendre les sites et les salariés du groupe dans les meilleures conditions possible. L’État, qui a déjà fourni un important soutien au groupe, continuera de l’accompagner dans ce contexte. Il veillera notamment à ce que les salariés bénéficient du meilleur accompagnement possible. Au delà de cette recherche de nouveaux partenaires industriels, le groupe est confronté à des facteurs exogènes qui menacent sa viabilité, ainsi que vous l’avez souligné. Ces facteurs tiennent notamment à un dépositionnement concurrentiel sur le sucre, qui constitue la principale matière première du groupe et que ce dernier est contraint d’acheter à des prix significativement supérieurs à ceux dont bénéficient ses concurrents extraeuropéens. En parallèle, le groupe subit sur sa production une concurrence très forte d’acteurs asiatiques, en particulier chinois. L’État L’État est pleinement mobilisé pour répondre à ces enjeux clés pour le groupe. Plusieurs pistes ont été identifiées et sont en cours d’examen pour soutenir la compétitivité du groupe, tout en le protégeant

L’usine d’Amiens a besoin de réponses rapides et d’un soutien sans faille pour atteindre ses objectifs, notamment garantir la souveraineté nationale dans l’approvisionnement des substances produites. La parole est à Mme Laurence Garnier,

L’éligibilité des dépenses est désormais effective lorsqu’elles sont imputées régulièrement sur un compte éligible figurant sur la liste fixée par l’arrêté interministériel modifié du 30 décembre 2020. À la suite de la concertation menée dans le cadre de l’Agenda territorial, et soucieux de poursuivre et d’amplifier son soutien à l’investissement des collectivités territoriales, territoriales, le Gouvernement a décidé que les dépenses d’agencement et d’aménagement de terrains seraient réintégrées dans l’assiette d’éligibilité au FCTVA, à compter du 1 janvier 2024. Du point de vue calendaire, conformément au code général des collectivités territoriales, ce fonds est liquidé par rapprochement entre les réalisations budgétaires d’un exercice et la liste des comptes éligibles au cours de ce même exercice, ainsi que le prévoit un arrêté interministériel. En d’autres termes, les droits au FCTVA sont déterminés au regard du cadre juridique applicable à date et ne peuvent donc faire l’objet d’un versement rétroactif.

L’extension rétroactive des dépenses d’aménagement de terrains entraînerait un coût évalué à près de 750 millions d’euros pour les exercices 2021, 2022 et 2023. Or le montant du FCTVA attribué est resté à des niveaux élevés au cours de cette même période. L’extension d’assiette est une mesure tournée vers l’avenir,

Cette restriction budgétaire est très inégalement répartie entre les dix programmes de la mission. Le programme 174, « Énergie, climat et après mines », concentre, à lui seul, plus d’un milliard d’euros d’annulation de crédits.

je souhaite que vous m’indiquiez quels sont les crédits alloués à la gestion économique et sociale de l’après mines, dont je crains qu’elle ne ressorte particulièrement lésée de la politique d’austérité de votre gouvernement. Je rappelle à votre mémoire le rapport pour avis du Sénat qui soulignait déjà le caractère peu protecteur du budget dévolu à la gestion de l’après mines du projet de loi de finances initiale Ces crédits doivent financer les dépenses sociales des anciens mineurs, mais aussi la dépollution du site Carling Saint Avold et les contentieux de Charbonnages de France. Nombreux sont les anciens mineurs victimes de maladies respiratoires et de cancers. Le tribunal de Metz croule sous les affaires de reconnaissance de maladies professionnelles ou de fautes inexcusables de l’employeur. Par ailleurs, le contentieux en cours relatif au déstockage du site du site StocaMine, en Alsace, est susceptible, à lui seul, d’accroître fortement les besoins de financement et de rendre insuffisant le calibrage de ces mesures budgétaires. L’annulation de crédits d’un budget déjà restreint n’aura t elle pas pour conséquence de pénaliser davantage la vie de ces anciens mineurs, qui luttent

deuxièmement, accompagner la transition énergétique ; troisièmement, accompagner la transition économique, sociale et environnementale des territoires touchés par des mutations industrielles liées à la transition énergétique. Il vise notamment à garantir aux anciens mineurs la préservation de leurs droits après l’arrêt de l’exploitation minière. En 2024, près de 90 % du programme 174, doté de 5 milliards d’euros, financent les trois principaux dispositifs d’aide versés aux ménages, à savoir la prime à la conversion des véhicules et le bonus écologique, le chèque énergie, dont l’objectif est d’aider les ménages à revenu modeste, la prime de transition énergétique dite MaPrimeRénov’.

aux communes. Depuis quelques années, le Gouvernement encourage et soutient la création volontaire de communes nouvelles, car ces structures permettent de maintenir une entité communale plus forte et vivante. L’État a acté l’idée d’un pacte financier pour sécuriser la commune nouvelle et faire en sorte que des communes qui se regroupent ne subissent pas de pertes financières.

de la dotation issue du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). En d’autres termes, ces communes perdent de l’argent, en tout cas des recettes qu’elles auraient pu

est à Mme la secrétaire d’État. Madame la sénatrice Gatel, le dispositif que vous citez, à savoir le fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité sur les mutations à titre onéreux, laisse effectivement au conseil départemental une assez grande liberté pour répartir ce fonds entre les communes de moins de 5 000 habitants, au titre de la libre administration des collectivités. Cette liberté est toutefois encadrée. D’une part, le barème doit prévoir trois critères : la population, les dépenses d’équipement brut et l’effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire. D’autre part, la répartition doit respecter le caractère péréquateur de ce fonds, c’est à dire contribuer à réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes. Il paraît difficile de regretter cette liberté confiée aux élus, qui est précisée par la loi. En outre, les conseils départementaux ont la possibilité de mettre en place des mécanismes de garantie pour certaines communes qui perdraient un montant trop important. Cette marge d’appréciation permet donc aux conseils départementaux, dans certaines conditions et s’ils le souhaitent, de garantir aux communes nouvelles tout ou partie du montant perçu par les communes préexistantes pour accompagner ces fusions de communes. En revanche, s’il est possible d’intégrer des mécanismes de garantie, ceux ci doivent être limités dans le temps et en volume financier, afin de ne pas remettre en cause le caractère péréquateur du fonds en entraînant

L’initiative, portée par le Gouvernement, consistant à mettre en place, en septembre 2023, une indemnité de résidence couvrant initialement 61, puis 133 communes situées près de la frontière suisse, dans les départements de l’Ain et de la Haute Savoie, est à saluer. Fixée à 3 % du salaire hors primes des agents publics bénéficiaires et représentant un montant annuel moyen avoisinant 840 euros brut, cette indemnité de résidence constitue à la fois un soutien financier et une reconnaissance pour les personnels des trois versants de la fonction publique qui y sont éligibles. Cependant, de nombreux agents publics travaillant dans d’autres départements, pourtant confrontés à des problématiques identiques, comme la fuite des compétences vers la Suisse, vers la Suisse, pays aux salaires bien plus attractifs, ou encore la flambée des prix de l’immobilier, source de bien des difficultés d’accès au logement, ne peuvent prétendre à ce dispositif. Face à cette situation, qui, loin d’être comprise par les acteurs sur le terrain, est même vécue comme une injustice, je souhaiterais connaître les raisons pour lesquelles le bénéfice de l’indemnité de résidence n’a pas été étendu à d’autres communes. Madame la secrétaire d’État, je vous demande donc si le Gouvernement envisage d’élargir prochainement ce dispositif à d’autres territoires frontaliers, notamment au département du Doubs,

est à Mme la secrétaire d’État. Madame la sénatrice Jacquemet, l’indemnité de résidence est calculée en fonction du lieu dans lequel les agents exercent leurs fonctions et du montant de leur rémunération. Plus précisément, l’indemnité de résidence est égale à un pourcentage de l’indice détenu par l’agent public. Le pourcentage varie en fonction de la commune : il est de 3 %, de 1 % ou nul, selon le classement de la commune ou de l’intercommunalité, comme j’ai eu l’occasion de le rappeler précédemment. Ce classement fait l’objet de mises à jour. Par exemple, au cours de la période récente, le décret du 12 décembre 2023 a permis aux agents exerçant dans 133 communes frontalières de l’Ain et de la Haute Savoie de bénéficier de l’indemnité de résidence à hauteur de 3 %. Au total, dans la fonction publique d’État, près de la moitié des agents

de résidence offre déjà un niveau de couverture important. Les demandes d’extension à d’autres communes doivent être examinées avec prudence, compte tenu de leur impact sur les finances publiques. Pour mémoire, en effet, le coût global de l’indemnité de résidence pour l’État s’élevait à près de 590 millions d’euros en 2023. Je l’ai dit, le député David Amiel s’est vu confier une mission sur ce sujet

est dans une situation alarmante. Nous avons pu constater de nombreuses infiltrations, moisissures, mais surtout l’effondrement partiel de murs ; les pignons de plusieurs bâtiments menacent de s’effondrer, contraignant la direction à prendre des mesures d’urgence. Une cinquantaine de détenus ont été transférés, la section des mineurs, fermée, de nombreuses cellules, désinfectées. Plusieurs lieux importants du parcours de réinsertion bibliothèque, foyer socioculturel, bureaux de l’éducation nationale, salle de sport, espace de formation professionnelle, ateliers de métallurgie – sont également fermés. La cuisine centrale est elle même désormais menacée.

Pour rappel, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme le 6 juillet 2023 pour violation des articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme. Si la situation des prisons en France pose de grandes difficultés, il y a, pour celle de Rouen, une urgence absolue. Il s’agit non plus de gérer les désordres au cas par cas, mais d’entreprendre une réhabilitation complète. Quelles mesures, madame la ministre, M. le garde des sceaux

Sans attendre, le ministère de la justice a décidé d’attribuer une enveloppe de 3,5 millions d’euros pour l’année 2024, afin que les opérations de maintenance les plus urgentes puissent être réalisées. être réalisées. Une opération de renforcement de certains murs pignons détériorés et d’éléments de la charpente en bois va effectivement être entreprise en priorité. Dans l’attente de l’achèvement du diagnostic du bâtiment, des mesures conservatoires seront mises en œuvre à court terme, afin, tout d’abord, de garantir la sécurité des personnes détenues et des personnels, ensuite, de mettre en place les prérequis à l’opération de renforcement structurel.

Les travaux de rénovation proprement dits concerneront en premier lieu la réfection complète de la couverture, le rejointoiement des façades en briques, le remplacement des menuiseries extérieures et la reprise intégrale des installations de plomberie sanitaire, de la ventilation et de l’électricité,

Vous le savez, monsieur le sénateur, les budgets de rénovation ont augmenté significativement, avec près de 140 millions d’euros par an depuis plus de cinq ans. Vous pouvez compter sur la mobilisation de M. le garde des sceaux pour poursuivre ces travaux.

et non d’une reconstruction, car cet établissement est idéalement situé, tant pour les personnels que pour les familles. Nous attendons donc des décisions plus importantes que celles que vous venez d’annoncer. La parole est

2 100 emplois ont été créés dans le cadre de la justice de proximité ; 700 magistrats et 850 greffiers supplémentaires ont également été recrutés. Ces premiers efforts se sont d’ailleurs traduits très concrètement pour nos concitoyens, avec une baisse significative des stocks d’affaires en cours de près de 30 %.

tiens, ici, à vous rassurer. Les départs de magistrats que vous évoquez et les vacances qui en découlent seront, dans la mesure du possible, compensés cette année par l’arrivée d’auditeurs de justice et de lauréats du concours complémentaire, doivent encore choisir leur poste. Depuis 2020, je le rappelle, 10 renforts sont arrivés au tribunal judiciaire du Havre dans le cadre de la mise en œuvre du plan Justice de proximité, dont 1 contractuel de catégorie A, 5 contractuels de catégorie B, 2 contractuels de catégorie C et 1 technicien informatique de proximité.

ont acté un projet de carte scolaire qui aboutira à la fermeture de 31 classes dans mon département du Cher pour la rentrée scolaire de 2024. Je pourrais, certes, critiquer les méthodes employées par le recteur ou le directeur académique des services ne font qu’appliquer une politique dont ils ne sont pas les instigateurs, une politique, je le regrette profondément, dictée par une logique comptable pure et dure. Cette logique comptable pèse lourdement sur nos maires, sur nos enseignants, sur les parents d’élèves et, inévitablement, sur nos enfants, réduisant nos écoles, nos classes à de simples statistiques : nombre d’élèves, taux d’encadrement, ratios, etc. tels indicateurs ignorent les efforts de nos municipalités et de nos instituteurs pour assurer un enseignement de qualité. Madame la ministre, je sais que Mme Belloubet a reçu des parlementaires du Cher de votre majorité pour discuter de ce sujet. Or, selon toute vraisemblance, la carte scolaire n’a pas tenu compte de leurs revendications. Nous savons également que des initiatives parlementaires ont été déposées à l’Assemblée nationale, mais, soyons réalistes, il y a peu de chances qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour.

Cette demande, je ne suis pas seul à la formuler : elle émane des élus locaux, des enseignants, des parents d’élèves et, plus largement, de tous ceux qui œuvrent au quotidien pour l’éducation de nos futurs citoyens. Il s’agit simplement de donner à ces acteurs du temps pour mieux s’organiser.

doit justement permettre de donner de la visibilité sur les perspectives à trois ans dans le premier degré. Nous suivons de très près les travaux de cette instance, au sujet de laquelle le ministère fera un point vers le mois de mai Des réponses adaptées aux territoires ruraux ont été élaborées au cours des dernières années : je pense notamment à l’allocation progressive des moyens, qui tient compte de l’indice d’éloignement, ou encore au dispositif Territoires éducatifs ruraux, au bénéfice des écoliers et des collégiens. insiste, la carte scolaire est le résultat d’un travail continu, pour s’adapter au mieux aux évolutions des effectifs scolaires. Or, dans le contexte regrettable de baisse démographique dans le Cher, dans le Cher, avec 2 683 élèves de moins, soit une baisse de 10 %, dans les écoles publiques du premier degré entre 2017 et 2023, et malgré les évolutions récentes de la carte, le taux d’encadrement dans votre département passé de 5,61 à la rentrée 2017 à 6,22 à la rentrée 2023, au dessus de la moyenne nationale, qui est de 6. Ce taux devrait encore augmenter à la rentrée prochaine. Je rappelle que le nombre d’élèves par classe était de 20 élèves à la rentrée 2023.

une expérience artistique dans le cadre d’un projet de classe. Cependant, la rentrée 2023 2024 a marqué un tournant, à la suite de deux mesures dont les effets de bord n’ont pas été anticipés. part, le ministère de l’éducation nationale a décidé de reporter la formation continue des professeurs hors du temps scolaire, ce qui a réduit leur disponibilité pour participer aux dispositifs d’éducation à l’image. part, les décrets des 8 et 9 août 2023 ont établi en parallèle de nouvelles obligations concernant les remplacements de courte durée (RCD), lesquelles ont contraint nombre d’enseignants à annuler les projections prévues avec les élèves. Ainsi, dans le premier comme dans le second degré, ces deux réformes ont véritablement fragilisé la politique d’éducation à l’image. Dans certains rectorats, le nombre d’élèves bénéficiant de cette initiation artistique a été divisé par deux.

Afin de ne pas répéter les erreurs commises, que prévoit le ministère pour concilier formation et présence des professeurs devant les classes et soutien à la politique d’éducation à l’image ? Qu’entend il mettre en œuvre pour garantir l’effectivité de ces dispositifs, qui, depuis tant d’années, ont fait leurs preuves ? La parole

En 2022 2023, quelque 55 % des élèves éligibles et 90 % des collèges et lycées ont profité du pass Culture. En 2023 2024, ces résultats seront largement dépassés. L’éducation au cinéma est l’un des piliers de l’éducation artistique et culturelle. Elle est le deuxième domaine d’utilisation de la part collective Madame la sénatrice, la mise en place du dispositif de remplacement de courte durée constitue également un enjeu majeur pour ce qui est des apprentissages – c’est le fond de votre question – et de la lutte contre les inégalités scolaires. Puisque nous avons décidé que les heures de formation ne devaient pas se faire au préjudice des élèves, l’enjeu est d’organiser les formations dans des conditions

Je ne veux pas opposer RCD et EAC. Nous travaillons donc à prendre en compte les contraintes des partenaires culturels, qui ne peuvent pas toujours accueillir les temps de formation sur ces temps d’ouverture au public que sont le mercredi après midi, le week end et les vacances. de faire en sorte que les chefs d’établissement disposent de la visibilité nécessaire sur les temps de formation, afin d’organiser au mieux les remplacements éventuels sur l’ensemble de l’année scolaire et, surtout, d’éviter que le report des temps de formation hors du temps scolaire ne soit source de démotivation pour les enseignants.

47 classes fermeront ; à Noyelles sur Mer, c’est l’école qui n’ouvrira pas ses portes à la rentrée prochaine. Si la mobilisation sans faille des élus, des syndicats,

le Gouvernement n’abandonne pas les territoires, la Somme en particulier, pas plus dans le domaine scolaire que s’agissant des autres politiques menées. Si nous devons adapter le service public de l’éducation à la réalité de la démographie de nos territoires, c’est bien pour assurer à tous les élèves les meilleures conditions d’enseignement.

en éducation prioritaire et limitation à 24 élèves en grande section de maternelle, CP et CE1, en préservant autant les zones rurales que les territoires urbains. Pour les collèges publics, à la rentrée 2024, les moyens d’enseignement sont maintenus dans la Somme, malgré la baisse prévue de centaines d’élèves, notamment collégiens. Les dotations globales horaires déléguées aux établissements doivent permettre un maintien des taux d’encadrement à la rentrée 2024, tout en accompagnant la mise en œuvre des mesures du « choc des savoirs », la poursuite de l’effort en faveur de l’école inclusive et les évolutions

Le remboursement des soutiens gorges compressifs, qui sont coûteux – de l’ordre de 100 euros par unité, et il en faut deux pour des raisons d’hygiène – n’est pas encore acté, alors que d’autres dispositifs comparables, en ce qu’ils participent à la reconstruction psychologique et physiologique des patients, le sont. À titre d’exemple, les ceintures de maintien abdominal, prescrites après une opération bariatrique, peuvent être entièrement remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle. De même encore, les perruques des patients ayant subi une chimiothérapie ou atteints d’alopécie sont désormais remboursées, ce qui met fin à une injustice. En effet, il était constaté que trop de malades y renonçaient pour des raisons financières. raisons financières. Ma question soulève également un problème de justice face à la maladie et d’équité de traitement. Le soutien gorge compressif est un complément indispensable à la reconstruction mammaire, à la suite d’un cancer du sein. La demande malheureusement existe, les fabricants la connaissent bien, mais ne soumettent pas de dossier à la Haute Autorité de santé (HAS), car la procédure est longue et coûteuse, et son sort aléatoire. Pour autant, l’inscription de ce dispositif sur la liste des produits et prestations remboursables pour les femmes ayant eu un cancer du sein, donc étant en affection de longue durée (ALD), est indispensable. Je souhaiterais vivement que vous me confirmiez que le Gouvernement l’envisage, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 par exemple. Au nom de toutes les femmes touchées et concernées,

générique de ce type de produit existe, le dispositif peut y être inscrit s’il respecte les exigences minimales requises décrites par un arrêté publié au. En l’absence de description générique, l’exploitant du dispositif peut également faire une démarche auprès de la Haute Autorité de santé, afin d’obtenir une inscription en nom de marque sur la liste. liste. L’inscription sur la liste conditionne la prise en charge par l’assurance maladie. Comme vous l’avez dit, madame la sénatrice, et cela me désole, aucun fabricant n’a formulé à ce jour de demande d’inscription pour ce type de dispositif, et il n’existe pas, actuellement, de ligne générique permettant leur prise en charge. De premières démarches d’industriels pour l’inscription peuvent être nécessaires, afin d’évaluer et de définir un cadre de prise en charge, avec des spécifications techniques, des indications ainsi que des modalités

L’État apporte alors une aide de 3 euros aux communes éligibles pendant trois ans. Les bénéfices de ce dispositif ne sont pas négligeables. Au delà de l’aide financière, la tarification sociale des cantines permet d’apprendre aux élèves de bonnes habitudes alimentaires et d’utiliser des produits un circuit court.

Cependant, des questions se posent quant aux modalités de la reconduction de la convention pluriannuelle entre l’État et les communes. Ainsi, les communes qui ont signé une telle convention en 2021 ne savent pas si le dispositif pourra être reconduit à compter de la rentrée de septembre 2024. Alors que les bénéfices de celui ci sont importants tant pour les communes que pour les élèves et leurs familles, je vous remercie de bien vouloir préciser si la convention pluriannuelle entre l’État et les communes mettant en place la tarification sociale des cantines sera reconductible, et selon quelles modalités. La parole est à Mme la ministre

et l’évolution de la mesure pour être en ordre de marche dès janvier 2024. Il est confirmé que les collectivités qui ont déjà une convention pluriannuelle peuvent la renouveler auprès de l’ASP au moment au moment de son échéance, sous réserve de continuer à respecter les critères d’éligibilité. Les collectivités qui le souhaitent peuvent signer à tout moment un avenant à la convention en cours pour bénéficier du bonus Égalim. Vous pouvez, monsieur le sénateur, compter sur la mobilisation du Gouvernement, notamment de la ministre Catherine Vautrin, qui est chargée des solidarités, pour poursuivre sur cette voie, parce qu’elle fonctionne

(AVA), ouverte à un plus grand nombre de bénéficiaires depuis le 1 septembre 2023. Il faut cependant continuer à travailler pour la reconnaissance et l’accompagnement des aidants. C’est pourquoi nous avons lancé, en octobre dernier, une nouvelle stratégie 2023 2027, élaborée en concertation

Grâce à cette possibilité, le temps d’attente aux urgences a baissé en moyenne d’une heure pour les patients présentant des symptômes grippaux et la prescription d’antibiotiques inutiles a été réduite. Les EBMD apportent des réponses immédiates et évitent surtout de multiplier les consultations. Ils contribuent donc au désengorgement du système de santé. Je voudrais rappeler l’historique : c’est à partir de 2014 qu’a été introduite la possibilité de confier la réalisation de ces prélèvements à un médecin non biologiste en dehors d’un laboratoire de biologie médicale. C’est dans la loi de financement de la sécurité sociale de 2020 que nous avons assoupli les règles pour garantir aux citoyens des services réactifs et sûrs.

Le Parlement a voté un modèle de financement pour les EBMD dans la loi de financement de sécurité sociale de 2023. Nous attendons donc les arrêtés de votre ministère pour que l’extension soit effective et légale,

relative à la biologie médicale. Initialement, elle permettait, uniquement pour une décision thérapeutique urgente, de réaliser la phase analytique d’un examen de biologie médicale en dehors du laboratoire de biologie médicale.

Le dispositif a de nouveau été modifié par la loi de financement de la sécurité sociale de 2023, qui prévoit son extension aux établissements médico sociaux et aux maisons de santé. La modification permet également aux agences régionales de santé de restreindre la biologie délocalisée aux seules structures éligibles au regard du contexte et des besoins territoriaux.

C’est ce qui est arrivé récemment au maire d’une commune de la Loire, qui, contacté par la famille d’une octogénaire dont elle n’avait aucune nouvelle, s’est rendu au domicile de cette dernière et l’a malheureusement découverte décédée, sans doute depuis plus de vingt

Loire – est difficile à vivre pour les personnes présentes sur place, pompiers, gendarmes et famille. C’est une conséquence rarement évoquée des déserts médicaux : il faut parfois plusieurs heures, lorsqu’un décès survient sur la voie publique ou au domicile, avant qu’un médecin ne puisse venir dresser un certificat, préalable indispensable à la levée du corps. C’est encore plus vrai lorsque le décès survient la nuit, durant les vacances ou lors d’un jour férié. Les Ehpad sont, eux aussi, confrontés à ce problème. Se trouve en cause, bien évidemment, la pénurie de médecins généralistes,

pourront établir un certificat de décès dans certains cas, moyennant le versement d’une indemnité. Aussi, face à de tels dysfonctionnements pérennes, notamment en zone rurale, pouvez vous me dire si le Gouvernement entend étendre rapidement l’expérimentation, conduite dans certains départements, qui permet à des infirmiers libéraux d’établir des certificats de décès ?

des solidarités. Madame la ministre, je me permets d’attirer votre attention sur l’un des aspects de la réforme du 100 % santé portant plus particulièrement sur les difficultés liées aux calculs et aux remboursements dans le secteur auditif. La réforme du 100 % santé a permis une avancée dans la prise en charge par la sécurité sociale des dispositifs optiques, dentaires ou encore auditifs. En effet, elle permet de supprimer le reste à charge sur les appareils de première catégorie, et cela doit être salué. Cependant, j’ai été alerté par un certain nombre de praticiens du département dont je suis l’élu, le Loiret, notamment des audioprothésistes, au sujet de la complexité et des incohérences dans les calculs de remboursement pour les appareils de seconde catégorie. En effet, une personne atteinte d’une affection de longue durée (ALD) et bénéficiant d’une prestation de compensation du handicap disposera d’un reste à charge plus important qu’une personne sans ALD. Par ailleurs, le secteur fait face à une augmentation très importante de la fraude principalement causée par l’usurpation d’identités et la réalisation de faux actes, ce qui est

Aujourd’hui, le collectif des infirmiers libéraux appelle à une journée de mobilisation dans toute la France. Mais ces infirmières et ces infirmiers manifestent déjà depuis plusieurs semaines dans de nombreux territoires, notamment dans ma région, l’Auvergne Rhône Alpes. Afin Afin de mieux comprendre leurs attentes, je suis allé à leur rencontre. Après quelques minutes de discussion, on comprend tout de suite que cette profession souhaite une meilleure reconnaissance et une amélioration de ses conditions de travail, qui, depuis de nombreuses années, évoluent vers une forme de précarité inquiétante. Pour illustrer cette évolution, prenons deux exemples. D’une part, les actes médicaux infirmiers, qui sont remboursés par la sécurité sociale, n’ont pas été revalorisés depuis 2009, autrement dit depuis quinze Pourtant, il n’aura échappé à personne que nous venons de traverser la crise inflationniste la plus importante depuis les années 1970, crise dont les effets se font encore ressentir. D’autre part, si les indemnités forfaitaires de déplacement ont été récemment revalorisées de 25 centimes, passant ainsi de 2,50 à 2,75 euros, force est de constater que cette augmentation est insuffisante aux yeux des professionnels. Compte tenu de l’inflation qui pèse sur les frais de fonctionnement d’un professionnel, les infirmiers libéraux travaillent en réalité pour un taux inférieur au Smic, si ce n’est à perte dans certains cas. Une telle situation n’est financièrement pas tenable pour la profession. Or ces infirmiers libéraux constituent un maillon essentiel de notre système de santé. Ils garantissent la continuité des soins et assurent un maillage territorial remarquable, notamment dans les zones les plus rurales de notre pays. Aussi, madame la ministre, pour que cette profession dévouée puisse perdurer, pour lui garantir une rémunération équitable et pour préserver l’accès aux soins de nos concitoyens, le Gouvernement peut il envisager, d’une part, la possibilité de revaloriser la tarification des actes médicaux infirmiers, et, d’autre part, une meilleure prise en compte de leurs frais de déplacement ? La parole

des patients dépendants en vue d’améliorer la qualité des soins, il représente un investissement de 714 millions d’euros pour l’assurance maladie. Nous devons achever la généralisation de ce mode de tarification à l’ensemble des patients dépendants.

des solidarités. Madame la ministre, ma question porte sur l’accès aux pratiques de soins intégratives et sur leur encadrement, demandé par les médecins thérapeutes eux mêmes.

vers des pratiques de soins non conventionnelles, et ce chiffre grimpe à 70 % chez les patients atteints de maladies chroniques, graves ou douloureuses. Depuis de nombreuses années déjà, nos voisins allemands et suisses, ainsi qu’une majorité de pays occidentaux, ont développé avec succès à l’hôpital ou en soins ambulatoires. En France, nos institutions entretiennent une confusion entre « bonnes » et « mauvaises » pratiques, au détriment des malades. Ceux qui le peuvent vont d’ailleurs se faire soigner à l’étranger.

en juin 2023, un comité d’appui technique à l’encadrement de ces pratiques, mais ses travaux sont à l’arrêt. Madame la ministre, quel est aujourd’hui le calendrier prévu pour avancer sur ce sujet ?

pourront s’envisager dès lors qu’une information objective fondée sur les résultats d’études scientifiques sera disponible. Le comité d’appui a permis de faire émerger un consensus parmi l’ensemble des

Pas plus tard que la semaine dernière, j’ai encore pu m’entretenir avec certaines d’entre elles. Toutes m’ont fait part de leur détresse, de l’absence de réponse à leur inquiétude et du désarroi dans lequel la fermeture du centre les a laissées. Cette situation met en péril la santé et le bien être de patients pourtant déjà vulnérables. Plusieurs d’entre eux se sont ainsi retrouvés en état d’acidocétose diabétique et ont dû être hospitalisés d’urgence. Si l’agence régionale de santé (ARS) se veut rassurante, notamment par la mise en place d’un numéro d’urgence, je ne puis que constater, sur le terrain, l’absence de solutions et les nombreux refus de prise en charge auxquels se heurte une grande majorité des familles. Alors que, dans le Haut Rhin, nous sommes proches de la Suisse et de l’Allemagne, l’urgence justifierait, pour les cas les plus graves, l’on y recherche des solutions. La détresse des parents et la nécessité de rétablir un lien de confiance entre eux et les autorités de santé plaident pour la mise en place d’un comité de suivi. rendre compte régulièrement de l’état d’avancement de la prise en charge des patients et identifier les obstacles que ceux ci rencontrent dans la continuité des soins. Par ailleurs, l’expérience de ce centre Edens met en lumière le besoin le besoin urgent d’une prise en charge locale adaptée, innovante et pluridisciplinaire du diabète pédiatrique, qui miserait sur les avancées technologiques dans le domaine médical. Aussi, madame la ministre, quelles mesures concrètes envisagez vous pour répondre à l’urgence remonter les anciens patients du centre Edens ? Êtes vous prête à entamer une réflexion sur les nouvelles modalités organisationnelles de prise en charge du diabète, pour répondre pleinement aux besoins constatés sur ce territoire ? La

qui a provoqué la fermeture du centre, plusieurs mesures locales ont été prises, parmi lesquelles la mise en place d’un numéro d’appel et l’organisation de modalités de restitution des dossiers médicaux. Grâce à votre mobilisation, madame la sénatrice, une réunion a été organisée le 7 mars dernier

qui a remis son travail en mars 2022 à la DHUP, afin que celle ci finalise le rapport. Depuis cette date, pour des raisons inconnues, le rapport n’a toujours pas été publié. D’abord annoncé pour la fin de l’année 2022, il a été ensuite repoussé au premier semestre 2023, puis à la fin de l’année 2023. Il est question désormais d’une publication au cours du premier trimestre 2024… Les professionnels de la sécurité incendie – industriels, sapeurs pompiers, assureurs – et les associations qui œuvrent régulièrement en faveur d’actions de prévention contre les incendies domestiques l’attendent pourtant, afin de pouvoir lancer de nouvelles actions de sensibilisation auprès de nos concitoyens. En effet, il a été démontré que les détecteurs de fumée sauvent des vies et permettent de limiter considérablement les dégâts matériels quand un début d’incendie est détecté à temps. Il serait d’autant plus opportun d’obtenir une publication dans les meilleurs délais que la plupart des détecteurs ou piles de détecteurs arrivent en fin de vie. En effet, d’une durée de vie approximative de dix ans, ces équipements ont été principalement achetés par les ménages entre le décret d’application de 2013 et la date d’objectif initial fixée en 2015. Ce document serait donc une occasion idéale pour communiquer sur la période de renouvellement nécessaire qui s’ouvre. Monsieur le ministre, êtes vous en mesure de nous indiquer une date ferme et définitive de publication d’un rapport attendu depuis bientôt trois ans ? Le Gouvernement entend il soutenir et accompagner des actions pédagogiques sur la prévention des accidents domestiques, comme cela avait été le cas au moment de la publication de la loi ? La parole

Martin, les dispositifs de détection de fumée sont rendus obligatoires par le code de la construction et de l’habitation dans l’ensemble des habitations individuelles ou collectives. L’objectif est double : détecter les fumées émises dès le début d’un incendie et émettre un signal sonore suffisant pour réveiller une personne endormie dans le logement où la détection a eu lieu. La loi Alur du 24 mars 2014 a modifié les obligations relatives à l’installation et à l’entretien des détecteurs, en les partageant entre le propriétaire bailleur et l’occupant du logement lorsque celui ci est loué. L’échéance d’entrée en vigueur de ces dispositions était fixée au 8 mars 2015. La mise en place des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée vise avant tout à réduire la mortalité liée aux incendies nocturnes. L’article 5 de la loi du 9 mars 2010 prévoit un rapport sur l’application et l’évaluation de ses dispositions. Ce document doit également rendre compte des actions d’information du public sur la prévention des incendies domestiques et sur la conduite à tenir en cas d’incendie qui ont été menées depuis la publication de cette loi. L’action du ministère s’est focalisée dans un premier temps sur les campagnes de sensibilisation et de communication destinées à accompagner les mesures de 2010, puis leur évolution de 2014.

Dans ce contexte, les services du ministère ont fait appel au Centre scientifique et technique du bâtiment, en raison de ses compétences en matière de sécurité incendie, afin de disposer d’éléments objectivés et consistants. Puisque vous m’interrogez à ce sujet, je serai très précis sur la date. Ces éléments sont en cours d’analyse et de concaténation. Je vous annonce que le rapport sera transmis au Parlement d’ici au 1 mai prochain. Le Gouvernement est particulièrement sensible aux enjeux relatifs à la sécurité incendie et aux actions mises en œuvre en la matière. Les détecteurs avertisseurs autonomes de fumée, et plus généralement les actions de prévention et de sensibilisation contre les incendies domestiques conduites par les acteurs, participent grandement à cet objectif de sécurité. Voilà, monsieur le sénateur, la date précise que je puis vous communiquer, en vous assurant de tout notre soutien et en saluant votre engagement sur le sujet. La parole est à Mme Sylvie Valente Le

Ces communes de taille modeste possèdent le plus souvent sur leur territoire un joyau patrimonial qui attire de nombreux visiteurs. C’est le cas par exemple de la commune de Pierrefonds, dans le département de l’Oise, dont le château, de renommée internationale, a été visité par 162 000 touristes l’an dernier. Cette affluence est impressionnante si on la rapporte aux quelque 2 000 habitants qui peuplent la commune. Or, si ces communes rurales servent de vitrine culturelle à notre pays et incarnent l’authenticité de nos terroirs, elles sont loin de profiter réellement de l’engouement touristique qu’elles suscitent. En effet, les retombées économiques liées à l’afflux de visiteurs reviennent principalement à d’autres entités. Ainsi, le produit de la taxe de séjour est capté par les offices de tourisme et les recettes suscitées par la visite des monuments qu’elles abritent échoient au Centre des monuments nationaux (CMN), qui en est le propriétaire. Pis encore, ces communes doivent supporter les charges supplémentaires qu’induit la venue massive de touristes : usure accélérée du mobilier urbain et de la voirie nécessité de mobiliser le personnel communal les week ends et les jours fériés. Pour Pierrefonds comme pour nombre d’autres communes réunies sous le label associatif Station verte, le tourisme est une aubaine économique et culturelle dont elles ne récoltent que trop peu les fruits. C’est d’autant plus vrai que, bien souvent, ces communes ne bénéficient ni du classement en commune touristique ou station de tourisme ni des avantages qui se rattachent à ces statuts, sans parler de de la baisse continue des dotations de l’État aux communes, facteur structurel de fragilisation des finances locales. Aussi, monsieur le ministre, comment envisagez vous de mieux répartir les gains économiques suscités par le tourisme dans les communes qui se trouvent dans une situation ingrate ? une situation ingrate ? Quels moyens avez vous l’intention de mettre en œuvre pour alléger les contraintes particulières pesant sur elles du fait de l’attrait touristique qu’elles suscitent

ou de résidences secondaires. Si leurs dépenses de fonctionnement sont supérieures à celles des autres communes, il en est de même des recettes de fonctionnement spécifiques, qui se caractérisent par leur dynamisme. L’une de ces recettes spécifiques est la taxe de séjour, dont le montant perçu en 2022 pour les communes touristiques s’élevait à 4 500 euros pour 100 habitants, contre moins de 500 euros pour les autres communes. Le produit total de la taxe de séjour était en forte hausse en 2022, de plus de 57 % par rapport à 2021. Il s’élevait à 190 millions d’euros pour l’ensemble des communes, hors Paris. Paris. Les communes incluses dans le zonage de la taxe annuelle sur les logements vacants ont également la possibilité de majorer de 60 % leur cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Enfin, les communes touristiques qui souhaitent investir peuvent également solliciter le soutien de l’État au travers de dotations d’investissement maintenues à un niveau élevé, comme la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) ou encore le fonds vert. Ainsi, quelque 1 138 opérations portées par des communes touristiques ont été financées par la DETR au cours de l’exercice 2022, pour un montant total de 63,8 millions d’euros, tandis que 617 projets ont été financés par la DSIL, pour un montant total de 110,5 millions d’euros. La commune de Pierrefonds, dans l’Oise, à laquelle vous faites référence, a par exemple bénéficié, entre 2018 et 2022, de plus de 220 000 euros de subventions au titre de la DETR et de la DSIL pour divers projets d’investissement, tels que la mise aux normes d’accessibilité des cheminements extérieurs du foyer Napoléon ou la création d’une réserve d’eau incendie. Elle a également bénéficié, en 2023, d’une subvention DETR de 67 500 euros pour aménager la rue de l’Armistice. Vous le voyez, madame la sénatrice, nous sommes à vos côtés pour développer l’ensemble de ces projets dans votre territoire et dans tous les territoires de France.

la délégation de compétence du conseil municipal au maire entraîne le dessaisissement du conseil municipal sur la matière concernée, ce qui rend toute délibération ultérieure non seulement superflue, mais également illégale pour cause d’incompétence. Or, paradoxalement, les services préfectoraux demandent désormais une délibération du conseil municipal pour valider l’adoption de l’opération et arrêter les modalités de son financement. Cette contradiction entre la lettre de la loi et les pratiques administratives instaure une incertitude préjudiciable pour les collectivités, pourtant désireuses de se conformer aux exigences réglementaires. Cette situation est d’autant plus problématique que des demandes de subventions avaient été précédemment acceptées sans délibération du conseil municipal. Or, bien qu’elles soient le résultat de cette délégation de pouvoir au maire, ces délégations requièrent la présentation de ces délibérations. Ce changement de pratique soulève des questions légitimes quant à l’accès des collectivités aux financements nécessaires à leurs projets. Face à cette situation, je sollicite de votre part, monsieur le ministre, des éclaircissements détaillés sur ces règles,

et ses modalités de financement ont été préalablement approuvées par le conseil municipal. La nécessité d’une délibération peut paraître une condition contraignante, et l’on peut en effet s’interroger à son sujet. Elle a toutefois pour objectif de s’assurer, premièrement, que le projet a bien été validé par le conseil municipal ou communautaire, et, deuxièmement, que son plan de financement a bien été prévu et approuvé par le conseil municipal. Cela permet de s’assurer de la viabilité des projets, donc d’éviter de perdre des crédits votés annuellement par le Parlement en les attribuant à des projets qui, hélas, ne verraient pas le jour.

Non seulement nous n’avons pas été suivis, mais le Gouvernement n’a malheureusement pas prévu non plus de mesures d’accompagnement pour les communes sortant de l’aire de revitalisation. Afin de ne pas fragiliser les initiatives locales mises en place dans ces territoires ex ZRR, il convient pourtant d’aider ces communes.

par le Sénat, après un an de concertation avec les parlementaires, les associations d’élus et les acteurs économiques et associatifs. Par ailleurs, je vous confirme que le Gouvernement porte une attention toute particulière aux communes sortantes. D’une part, D’une part, il n’y aura pas de sortie sèche : les entreprises et professions médicales profitant actuellement des exonérations continueront à en bénéficier jusqu’à la date initialement prévue, jusqu’à extinction de leurs droits. D’autre part, je vous confirme que ces communes font d’ores et déjà l’objet d’un accompagnement spécifique. Ainsi, comme les parlementaires et élus locaux qui m’ont saisi le savent, toutes les mesures du plan France Ruralités seront activées en fonction des besoins de chaque territoire. Le zonage FRR constitue en effet un seul des quatre axes de France Ruralités. Ainsi, les chefs de projet Villages d’avenir, en plus de Petites Villes de demain, et les volontaires territoriaux en administration (VTA) sont à disposition des territoires. Les crédits d’ingénierie, considérablement augmentés dans la loi de finances pour 2024, seront également mobilisés en priorité

Par ailleurs, si nous sommes vigilants sur les communes touchées par un effet de seuil, maintenir de façon artificielle dans le dispositif les 2 400 communes sortantes, comme cela a été fait en 2015, ne ferait malheureusement que fragiliser les 4 000 communes

remercie, monsieur le ministre, de votre réponse. Soutenir les communes exclues des ZRR et les accompagner le temps de redresser la situation de manière non précipitée me semble important.

des territoires. Monsieur le ministre, les coupes rases en forêt font l’objet de controverses particulièrement fortes ces dernières semaines. Des associations alertent sur leur multiplication et leur impact. Plusieurs médias ont traité le sujet à des heures de grande audience et des riverains sont allés jusqu’à bloquer des chantiers. Les demandes d’encadrement font suite à la publication de l’expertise CRREF commandée par le ministère auquel vous êtes rattaché et par le ministère de l’agriculture. Cette expertise souligne notamment les effets néfastes de ces pratiques pour les sols et le microclimat forestier. Elle indique également que plus les coupes rases sont grandes, plus l’impact sur la biodiversité est élevé. Étant donné que le puits de carbone en forêt française a été divisé par deux au cours des dix dernières années et que 27 % des espèces forestières françaises sont menacées ou quasi menacées selon il apparaît en effet prioritaire d’encadrer les coupes rases et de mettre en avant la sylviculture mélangée à couvert continu. Cette pratique permet de récolter du bois de qualité en alliant les enjeux économiques et environnementaux. Deux propositions de loi récemment déposées à l’Assemblée nationale envisagent des mesures en ce sens. Le Président de la République a annoncé vouloir planter un milliard d’arbres d’ici à 2032 pour faire face au changement climatique. Au delà de l’effet de communication, c’est une véritable politique d’adaptation des forêts qui doit être bâtie avec tous les acteurs. Monsieur le ministre, le règlement européen sur la restauration de la nature a été adopté le 27 février Comment comptez vous appliquer ce règlement, notamment en matière de restauration des écosystèmes forestiers ? Soutenez vous les textes déposés dernièrement pour encadrer les coupes rases

Le débat se focalise trop souvent, à mon sens, sur les coupes rases. La surface de forêt hexagonale a doublé depuis le milieu du XIX siècle, et le volume de bois sur pied a augmenté de plus de 50 depuis les années 1980. Les indicateurs de bois mort et de diversité des essences recensés par l’IGN progressent depuis vingt ans, signe d’une biodiversité mieux préservée en forêt que dans d’autres milieux. Cependant, un réchauffement de 2,5 à 3,5 degrés Celsius à l’horizon 2050 aura des effets majeurs sur les forêts françaises. Trois priorités fondent notre stratégie d’adaptation forestière d’abord, accompagner nos forêts vers de nouveaux profils sylvicoles, avec des bouquets d’essences diversifiées et adaptées au climat sec et chaud ; ensuite, valoriser en usage matériaux les bois actuellement présents dans nos forêts avant que leur qualité technologique ne se dégrade au point de les condamner à un usage bois énergie ; enfin, étendre et amplifier la prévention des incendies. Ces priorités figurent en bonne place parmi les objectifs du prochain plan national d’adaptation au changement climatique qui sera soumis à la consultation du public par le ministre Christophe Béchu dans les prochaines semaines. La transition forestière nécessitera agilité et innovation. Elle passera par une diversité de solutions et de modes de sylviculture adaptés au profil des peuplements forestiers, qu’au contexte de chaque massif, loin des idéologies, des carcans et d’un modèle unique dans lesquels certains souhaiteraient enfermer les propriétaires forestiers. La transition forestière oblige à être encore plus attentif aux enjeux de la protection du capital naturel que constituent les sols forestiers et la biodiversité et à renforcer le mélange des essences de reboisement. Les propositions de loi que vous avez évoquées contiennent effectivement des mesures qui vont en ce sens. Il reviendra au Parlement de se prononcer à leur sujet. La transition forestière appelle surtout à l’action, à une mobilisation collective et positive aux côtés de ceux qui sont en première ligne face au défi du changement climatique. Je pense aux propriétaires, aux gestionnaires, aux exploitants et aux industriels du secteur forestier.

de Paris 2024. Cette décision aura un impact significatif non seulement sur eux, mais également sur les usagers de ces moyens de mobilité. Pour résumer, ces hommes et des femmes qui n’ont rien – ni droit ni protection

il devient impératif de garantir des conditions de travail décentes pour les conducteurs de VTC. C’est d’ailleurs le sens de la directive européenne qui vient d’être adoptée sur les droits des travailleurs des plateformes. Dans cette perspective, monsieur le ministre, quelles sont les mesures que le Gouvernement compte mettre en place afin d’éviter que les chauffeurs de VTC ne soient VTC ne soient exclus lors des jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris à partir de juillet 2024

non les VTC –, sous réserve de la fluidité du trafic et à l’appréciation du préfet de police. Pour la plupart, une seule voie est mobilisée sur l’axe routier, les autres voies restant, bien entendu, accessibles à l’ensemble des usagers.

Par ailleurs, les clients des VTC pourront accéder aux différentes zones ouvertes à la circulation sur le territoire francilien. Les chauffeurs VTC ne seront ni pénalisés ni exclus des jeux Olympiques 2024. Nous avons besoin de la mobilisation de tous les opérateurs de mobilité

bénéficient d’une équivalence. Les chauffeurs indépendants de VTC sont, par ailleurs, soumis à des règles d’accès à la profession : inscription sur un registre, honorabilité, garantie financière… Le Gouvernement a mis en place, sous l’égide de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi en place, depuis 2021, les premiers accords entre les plateformes et les chauffeurs visant à la régulation sociale du secteur. Je pense, par exemple, aux règles applicables par les plateformes en cas de désactivation des comptes ou à la mise en place d’un revenu minimal par course. a réaffirmé, par ordonnance, les principes d’indépendance qui doivent prévaloir dans la relation entre les plateformes et les travailleurs. Cependant, le Gouvernement reste vigilant sur la pérennité et l’équilibre de ce dialogue.

des territoires. Monsieur le ministre, la loi du 27 décembre 2019 permet aux communautés de communes de déléguer, par convention, tout ou partie des compétences eau, assainissement et gestion des eaux pluviales urbaines à une commune ou à un syndicat infracommunautaire existant au 1 janvier 2019. Des communes exercent actuellement la compétence « eau ». Elles assurent, des conventions, la production par captage puis la fourniture d’eau potable pour plusieurs autres. C’est, par exemple, le cas de la commune de Villelongue, dans les Hautes Pyrénées, qui, grâce à six sources captées, assure la fourniture d’eau potable pour ses habitants et ceux de trois autres communes voisines, soit 2 070 habitants au total. Ces conditions d’organisation de distribution d’eau potable sont régies par des conventions entre les communes

pourront perdurer par conventionnement avec l’intercommunalité au delà de cette date l’accès à l’eau potable représente un enjeu fondamental sur l’ensemble du territoire national. L’échelon communautaire a été choisi par le législateur pour remédier aux difficultés sanitaires, économiques et écologiques engendrées par l’émiettement des services. En effet, la mutualisation des moyens financiers et d’expertise à cette échelle permet d’améliorer la résilience et de moderniser les réseaux de distribution d’eau potable. C’est cette logique qui sous tend le transfert obligatoire aux communautés de communes de la compétence eau au 1 janvier 2026. Concrètement, cela signifie que l’ensemble des composantes du service d’eau potable, de la production à la distribution, en passant par le transport et le stockage, sera assuré par les communautés de communes. En conséquence conséquence de ce transfert, la communauté de communes se substituera de plein droit aux communes qui la composent dans tous leurs actes, dont les éventuelles conventions concernant la production et la fourniture d’eau potable. Toutefois, madame la sénatrice, je tiens

chargé des transports. Monsieur le ministre, les aéroports régionaux et les lignes d’aménagement du territoire (LAT) traversent aujourd’hui des zones de turbulence. Depuis 2002, l’État a mis en place des obligations de service public (OSP) sur des liaisons aériennes métropolitaines, afin que puissent être desservies des destinations qui ne le seraient pas dans les conditions normales du marché. Ces territoires sont également desservis de manière catastrophique par le réseau ferré.

PGE. Que s’est il passé depuis cette date ? En guise de remerciement envers la Nation, Air France a abandonné tous les territoires ruraux les uns après les autres lors des renouvellements des OSP. L’entreprise ne fait même plus acte désengagement fut l’aéroport de Brive, dans mon département, puis ce fut le tour de tous les aéroports, à chaque renouvellement d’OSP. Par exemple, Air France a abandonné Rodez, Aurillac, Limoges, Le Puy en

ma question est simple : allez vous demander à Air France de réviser sa position et de reprendre ces lignes d’aménagement du territoire, soit en direct, soit en affrètement, comme il le faisait dans de nombreux aéroports avant cet abandon tragique ? La parole est à M. le ministre délégué.

Depuis la crise sanitaire, le trafic aérien en métropole a connu des évolutions structurelles, en raison notamment des changements des habitudes de travail. On observe une diminution très sensible du trafic lié aux voyages d’affaires : le nombre de passagers faisant des allers retours dans la journée a baissé de 60 %. Tandis qu’en novembre 2023, le trafic aérien, en France, dans son ensemble, avait rejoint son niveau de 2019, le trafic domestique dépassait à peine 75 % de son niveau d’avant la crise. Ce contexte a bien évidemment bouleversé l’équilibre économique de toutes les lignes d’aménagement du territoire. La baisse constatée du trafic et l’augmentation de certains postes de coûts ont provoqué une augmentation des compensations financières demandées aux collectivités locales et à l’État. Face à la hausse de ces compensations, certaines collectivités ont fait le choix de supprimer la délégation de service public, d’autres de réduire le service. Le groupe Air France, qui exploitait quatre lignes d’aménagement du territoire avant la crise sanitaire, a tenu son engagement de ne pas dénoncer les délégations de service public en cours. Malgré les pertes, Air France et HOP ! ont ainsi été contraints d’aller jusqu’au terme de l’exécution des conventions de délégation de service public. Dans le même temps, Air France doit mettre en œuvre toutes les solutions permettant de mettre fin aux pertes rencontrées sur le réseau domestique, ce qui explique le désengagement progressif des LAT entrepris par la compagnie. Face à cette réalité, l’État demeure aux côtés des collectivités qui renouvellent et financent les contrats de délégation de service public. En 2023, 22 millions d’euros y ont été consacrés, dont plus de la moitié pour les LAT métropolitaines. Outre ces montants, l’État apporte également toute son aide technique aux collectivités pour la définition d’obligations de service public qui soient le mieux ajustées possible pour répondre à la défaillance du marché,

le trafic a été plafonné depuis 1994. Malheureusement, cet aéroport s’est étendu sur quatre îlots, et ce sont maintenant plus de 740 000 riverains qui subissent l’augmentation du trafic aérien, avec une exposition au bruit qui, bien évidemment, a des conséquences directes sur leur santé.

de l’aéroport d’Orly à celui de la métropole du Grand Paris, qui a été voté à l’unanimité des 131 communes membres. Aussi, monsieur le ministre, ma question est elle simple : le Gouvernement a t il l’intention de prendre cette mesure pour faire en sorte que les riverains aient enfin sept heures consécutives pour dormir, ce qui serait bon pour leur santé ?

et, depuis 1994, le trafic y est plafonné à 250 000 créneaux par an. Le plan de prévention du bruit dans l’environnement de l’aéroport, qui a été approuvé le 17 mars 2022, prévoyait la réalisation d’une étude d’impact selon l’approche équilibrée, sur laquelle les ministres chargés de l’environnement et des transports pourraient s’appuyer pour adopter de nouvelles restrictions d’exploitation. Le plan de prévention prévoyait de diminuer le bruit généré entre vingt deux heures et six heures d’au moins 6 décibels par rapport à la situation de référence de 2018 et, sur le même périmètre, de diviser par deux l’indicateur sanitaire de fortes perturbations du sommeil. Ces objectifs du plan de prévention ont été pris en compte dans l’étude d’impact dirigée par la préfète du Val de Marne. Toutefois, cette étude a mis en évidence un biais dans l’indicateur acoustique retenu de nature à fragiliser l’objectif de réduction du bruit de 6 décibels contenu dans le PPBE. Ce constat a été partagé avec l’ensemble des parties prenantes, dont les élus locaux concernés, lors d’une réunion d’information qui s’est tenue le 26 octobre 2023. L’étude d’impact est maintenant finalisée, et plusieurs scénarios de restriction ont été soigneusement étudiés. Ils comportent chacun des mesures ambitieuses, d’un niveau inédit Monsieur le sénateur, soyez assuré que le ministre de la transition écologique et le ministre chargé des transports tireront prochainement de ces travaux toutes les conclusions utiles à la préservation de l’équilibre entre les intérêts économiques des territoires, d’une part, et la protection de la population contre les nuisances sonores, d’autre part. Je vous confirme, enfin, sur un plan plus général,

Dans ce cadre, les décisions d’admission en non valeur peuvent être déléguées par l’organe délibérant à l’exécutif local. Cependant, c’est au pouvoir réglementaire qu’a été laissé le soin de fixer le seuil de ces montants : le décret du 29 juin 2023 a ainsi fixé ce seuil, pour les communes, à 100

pour les services administratifs de nos mairies. Dans le cadre de la démarche de simplification de l’action publique locale annoncée, je vous sollicite afin que les conseils municipaux puissent fixer eux mêmes un montant maximal des créances irrécouvrables au delà duquel une telle délégation ne peut advenir, au même titre que pour d’autres délégations, comme l’avaient prévu les parlementaires. moi, monsieur le ministre, d’insister sur la nécessaire reconnaissance de la libre administration de nos collectivités par des hommes et des femmes qui ne ménagent pas leur peine au quotidien. Comme je vous ai sous la main, je poursuis au delà de ma question… Nous sommes très souvent interpellés par les maires et les acteurs économiques locaux sur les enjeux de votre prochain projet de loi sur le logement.

des créances irrécouvrables de faible montant, l’article 173 de la loi 3DS ouvre la possibilité aux assemblées délibérantes des communes, départements et régions de déléguer cette décision à leur exécutif. La détermination du seuil plafond de délégation des décisions d’admission en non valeur a pour objectif de garantir la sincérité comptable, en admettant plus rapidement en non valeur l’ensemble des créances irrécouvrables, tout en garantissant aux assemblées délibérantes la maîtrise des impacts budgétaires. Ce seuil, fixé par le Gouvernement, a été défini conjointement avec les associations d’élus, afin de garantir un équilibre satisfaisant pour l’ensemble des acteurs de la chaîne de recettes.

des territoires. Monsieur le ministre, le décret n° 2019 461 et l’arrêté du 7 août 2019 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation interdisent désormais l’emploi de bardage bois en cas de rénovation de façades pour les constructions de 28 mètres, et de 9 mètres lorsqu’il s’agit d’un établissement recevant du public. Dans les stations de sports d’hiver, la majorité des constructions sont en bois et sont donc concernées par cette nouvelle réglementation, qui va à l’encontre non seulement de l’aspect architectural originel des stations et de l’identité de montagne, mais aussi de la filière bois française et des exigences d’une rénovation thermique écologique et efficace. En Haute Savoie, la commune de Morzine, labellisée « Patrimoine du XX siècle » et « Architecture contemporaine remarquable », est particulièrement inquiète des conséquences, pour son patrimoine, de ces nouvelles règles, qui imposent l’usage de matériaux composites, d’aluminium ou de plastique. Les communes hautes savoyardes de La Clusaz, Châtel ou encore Les Gets sont elles aussi concernées, et, dans l’ensemble, toutes les stations du territoire français pourraient être pénalisées. Aussi, monsieur le ministre, je souhaite savoir s’il serait envisageable de prévoir un moratoire sur l’application de cette réglementation,

dont la commune de Morzine Avoriaz est le parfait exemple. La réglementation relative à la sécurité incendie a été mise à jour en 2019 pour ce qui concerne les dispositions applicables lors de la rénovation des façades des bâtiments existants. Celle ci définit des critères quant à la réaction aux feux de façades, avec une exigence croissante en fonction de la hauteur du bâtiment. Elle fait notamment suite à l’incendie de la tour Grenfell, au Royaume Uni, dont la propagation très rapide a été attribuée à la présence du matériau d’isolation installé lors de la rénovation de la façade de l’immeuble. Plus récemment, l’incendie mortel d’un immeuble d’habitation à Valence, en Espagne, attribué à l’isolant, s’est également propagé par la façade. Les façades sont façade. Les façades sont un point d’attention majeur de la sécurité incendie, car elles permettent la propagation rapide du feu aux étages supérieurs et aux bâtiments situés à proximité. Les évolutions réglementaires se sont appuyées sur une recommandation du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB). Elles visent à prévenir de tels événements et à garantir la sécurité des occupants. Le Gouvernement considère que la sécurité des occupants est une priorité et n’envisage donc pas de revoir à la baisse les exigences de cette réglementation ou d’y ajouter de nouvelles dérogations. En revanche, il est important de rappeler que la réglementation permet de recourir à une approche alternative. Ainsi, sous réserve d’études spécifiques demandées à un laboratoire agréé en réaction et en résistance au feu, il est possible de faire valider une solution constructive innovante permettant d’utiliser du bois, sous certaines conditions techniques à définir. Si la performance d’un bardage bois au regard de la sécurité incendie est reconnue par le laboratoire, les exigences réglementaires pourront être satisfaites. J’invite donc les communes et les acteurs qui souhaiteraient adopter cette approche alternative

des territoires. Monsieur le ministre, pour créer légalement un projet d’autoconsommation collective étendue, le point de soutirage et le point d’injection des participants ne peuvent être séparés que par une distance maximale de 2

aller jusqu’à 20 kilomètres entre les participants. La méthode était souple, avec un dialogue constructif entre l’État et les territoires. Malheureusement, depuis l’arrêté du 19 septembre 2023, ce n’est plus possible. Désormais, pour que l’on puisse espérer une dérogation, il faut que le lieu du projet soit classé exclusivement sur une ou plusieurs communes rurales au sens de

Avant la modification, le Sdis pouvait obtenir dix dérogations. Après la modification, seules quatre zones se conforment aux nouveaux critères. Concrètement, c’est le projet de tout un territoire, et potentiellement celui des sapeurs pompiers, qui est Monsieur le ministre, je vais aller à l’essentiel et faire simple : il faut changer l’arrêté. Le Sdis de l’Isère, c’est 85 000 interventions, 112 casernes, 5 300 agents, 6 000 mégawattheures par an. Grâce à ce projet, ce Sdis espérait diminuer de 20 % sa consommation sur le réseau, réduire sa facture

et développer l’intervention d’urgence. En responsabilité, nous ne pouvons pas faire d’économies sur le dos de nos sapeurs pompiers ! Sans la modification de l’arrêté, le projet échouera, car c’est sa viabilité, rien de moins, qui sera remise en cause. Monsieur le ministre, il faut laisser nos territoires entreprendre et développer les énergies renouvelables décarbonées. Nous avons des objectifs nationaux à atteindre. Dès lors, soyons pragmatiques ! Pouvez vous vous engager à modifier cet arrêté ? La parole est à M. le ministre

Des dérogations à ce critère de proximité géographique peuvent être accordées sur demande motivée auprès du ministre chargé de l’énergie. Depuis 2020, la distance maximale peut ainsi être étendue jusqu’à 20 kilomètres pour les projets situés en zone rurale ; depuis 2023, elle peut atteindre jusqu’à 10 pour les projets situés en zone périurbaine. Cette dernière évolution n’a pas rendu les critères précédents plus contraignants : au contraire, elle a apporté une base légale plus solide pour justifier les décisions, en complétant les possibilités de dérogation et en en prévoyant une nouvelle, de 10 kilomètres au maximum,

aux critères prévus. Au risque de vous décevoir, monsieur le sénateur, il n’est donc pas exact d’affirmer que l’arrêté du 19 septembre 2023 a fait échouer ce projet. Je vous rappelle, enfin, que, l’autoconsommation étant un modèle dérogatoire et simplifié de fourniture,

Les contraintes que nous rencontrons sur le terrain, en particulier dans les zones rurales, comme celles de mon département, nous amènent à nous interroger sur l’adaptabilité de la loi à la diversité des situations locales.

À cela s’ajoute un contexte hydraulique qui complexifie les projets de rénovation de voiries. Il existe ainsi des accotements enherbés qui pourraient, s’ils étaient aménagés, répondre aux obligations de prise en compte du cyclable et des piétons.

à leur encontre ? Une telle flexibilité est essentielle pour permettre une adaptation plus fine aux spécificités locales, tout en respectant les objectifs environnementaux et de mobilité durable.

La loi d’orientation des mobilités de 2019 a étendu les possibilités d’aménagements pour répondre à cette obligation : bandes cyclables, voies vertes, zones de rencontre, etc. Depuis, ces différentes formes d’aménagements offrent aux collectivités un éventail de solutions pour répondre aux besoins des cyclistes, tout en tenant compte des contraintes que vous venez d’évoquer. dans la majorité des cas, il est possible, en agglomération, de réaliser ces aménagements sans extension de l’emprise de la chaussée. Lorsque ces aménagements sont réalisés à l’occasion de travaux programmés, le surcoût est limité – c’est la raison d’être de cette disposition. Les collectivités peuvent s’appuyer sur les recommandations

Ces centres offrent des services aux familles et aux habitants de proximité. Ils contribuent à la cohésion sociale dans les territoires, en renforçant le pouvoir d’agir des familles et des habitants, ainsi qu’en facilitant l’accès aux droits.

Ces ambitions et ces engagements ont été nourris par les bilans annuels des actions de la COG précédente, par les rapports d’évaluation de l’inspection générale des affaires sociales et par les besoins exprimés par les représentants des structures, partenaires locaux et nationaux des caisses d’allocations familiales. De surcroît, la COG prévoit un soutien financier à la création de 611 nouvelles structures, dont 150 centres sociaux et 461 espaces d’animation de la vie sociale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ainsi que dans les zones de revitalisation rurale les territoires non couverts. Ces mesures de rééquilibrage territorial ont pour ambition d’apporter un soutien à toutes les familles, et plus particulièrement aux plus précaires d’entre elles, qui disposent d’un moindre accès à leurs droits et aux services en soutien à la parentalité. Le but est de favoriser le maillage des structures d’animation de la vie sociale, en ciblant les territoires faiblement couverts. À titre d’illustration, la création de 50 centres sociaux supplémentaires a été intégrée, en juillet 2023, en comité interministériel des outre mer, aux 72 mesures concrètes pour améliorer le quotidien des Ultramarins. Ce soutien affirmé à la stratégie de développement des centres sociaux traduit, plus largement, l’engagement fort du Gouvernement à sécuriser et à pérenniser le fonctionnement des structures d’animation de la vie sociale, dans le contexte inflationniste actuel. Une revalorisation des prestations de services, des animations collectives destinées aux familles et des animations locales est prévue, afin de soutenir les salaires les salaires des professionnels de ces structures. Par rapport à la précédente COG, 80 millions d’euros supplémentaires seront dédiés au fonctionnement desdits centres. Le Gouvernement a néanmoins conscience des difficultés actuelles qui affectent un certain nombre de centres sociaux, fortement impactés par l’inflation et par la croissance de la demande sociale. La ministre du travail, de la santé et des solidarités rencontrera prochainement des représentants du bloc communal pour évoquer cette question. La possibilité d’un nouveau soutien d’urgence à destination des centres les plus fragilisés est également à l’examen. La parole

La séance est suspendue.